spéciale ? Ces deux amendements tendent à supprimer l'article 1 du projet de loi, qui prévoit un allégement de formalisme et la suppression de l'interdiction de certaines mentions dans les publicités relatives aux crédits à la consommation. Comme lors de l'examen du texte en commission, j'y suis défavorable, car j'approuve globalement ces simplifications en matière de droit de la consommation, qui répondent à une demande des entreprises, s'agissant de cas de surtranspositions avérés, et qui représentent, somme toute, des modifications mineures. En premier lieu, les trois dispositions que prévoit de modifier l'article 1 ne sont aucunement exigées par la directive de 2008 relative aux contrats de crédit à la consommation. Il s'agit donc bien de surtranspositions. En deuxième lieu, les modifications proposées dans le projet de loi sont très légères : le changement de taille de police de caractères ou la suppression d'un encadré n'emporteraient aucune déperdition d'information pour le consommateur, puisque les mêmes informations seraient toujours mentionnées sur les publicités. Les informations essentielles sur le coût du crédit resteront bien incluses dans toutes les publicités, quel qu'en soit le support. De plus, il n'est pas avéré que les dispositions actuelles aient un quelconque effet sur le comportement du consommateur en matière d'appréhension du risque. Enfin, s'agissant de l'interdiction de la mention dans une publicité de l'existence d'un remboursement différé, j'estime qu'il n'y a aucune raison de la maintenir, puisque ce remboursement ne constitue pas une offre illicite ; il s'agit en outre d'informer le consommateur. En troisième lieu, si j'estime bien évidemment que les mesures prévues à l'article 1 ne sont pas suffisantes, je ne vois pas de raison de m'y opposer. En effet, elles constituent un premier pas dans la dé-surtransposition et correspondent à une attente des entreprises, qui nous l'ont confirmé lorsque nous les avons entendues. Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable sur les amendements identiques n pour les mêmes raisons que le rapporteur. Les obligations imposées aux annonceurs que le Gouvernement propose de supprimer, outre qu'elles vont effectivement au-delà des exigences fixées par la directive, n'ont en réalité aucune valeur ajoutée en termes de protection des consommateurs- une protection qui reste une priorité du Gouvernement. Elles constituent dans le même temps des contraintes pour les entreprises. Concernant la taille des caractères dans lesquels doivent figurer certaines mentions obligatoires, le projet de loi rétablit la situation antérieure à la transposition de la directive de 2008 en prévoyant que ces informations peuvent figurer dans une taille au moins aussi importante que les autres informations. Il permet un assouplissement des contraintes des professionnels en matière de conception et d'édition des publicités, tout en garantissant que les informations non essentielles ne seront pas indûment mises en valeur par rapport aux informations essentielles. Quant à l'encadré, sa présence n'apporte aucune information supplémentaire aux consommateurs : il s'agit simplement d'une répétition, sous une autre forme, d'informations figurant déjà dans la publicité, de manière visible et lisible, conformément aux prescriptions de la directive. Au surplus, le consommateur disposera à nouveau de ces informations avant de contracter avec le prêteur dans la fiche d'information précontractuelle qui lui est obligatoirement remise.

Depuis la loi de juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, nous avons pu observer que ces dégâts étaient de plus en plus limités, parce

à convaincre un certain nombre de personnes qui pouvaient être facilement entraînées de faire plus attention. Il est donc important, utile et nécessaire de maintenir les dispositions dont la suppression

Ne pas voter ces amendements, approuver l'article 1, sur un premier texte destiné à régulariser ce que l'on appelle les surtranspositions de directive, serait donner un mauvais signe à la protection des consommateurs.

par les services financiers, mais obtenus par les démarches volontaristes et les revendications des consommateurs et, peut-être, d'un certain nombre de responsables politiques qui pensent à les protéger.

n° 8. L'article 1 , introduit en commission spéciale, supprime l'obligation faite aux prêteurs en matière de crédit renouvelable de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans.

à ces offres de crédit, avec des souscriptions qui peuvent paraître très alléchantes mais, finalement, participent au phénomène de surendettement. Alors que les personnes surendettées ont très souvent un ou plusieurs crédits renouvelables associés à une ou plusieurs cartes

se surendetter sans dispositif de prévention qu'on rendra notre économie plus dynamique ? Je ne suis pas convaincu que ce soit la piste d'avenir pour un pays comme la France.

et 30 rectifié tendent à supprimer l'article 1 , introduit par la commission spéciale, qui abroge l'obligation faite aux prêteurs en matière de crédit renouvelable à la consommation de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans. Cette obligation constitue pourtant une surtransposition qui a un vrai coût pour les entreprises, qui nous l'ont d'ailleurs signalé en audition. Il s'agit d'une vraie mesure de fond, que j'ai proposée et sur laquelle la commission spéciale m'a suivi. En premier lieu, cette obligation de vérification triennale constitue une surtransposition de la directive relative aux contrats de crédit au consommateur. Le droit de l'Union européenne n'impose en effet la vérification de la solvabilité de l'emprunteur qu'en amont de la conclusion du contrat et avant toute augmentation significative du montant du crédit. Cette surtransposition a d'ailleurs été identifiée par la mission inter-inspections

suscitant des incompréhensions chez les emprunteurs, qui, souvent, ne sont pas coopératifs. En deuxième lieu, un contrôle est obligatoire également au cours du contrat de crédit, l'application des règles de détection précoce des risques d'insolvabilité et de fragilité des emprunteurs.

La loi de 2010 a renforcé l'examen de la solvabilité en exigeant non seulement cette vérification, mais aussi qu'elle repose sur un nombre suffisant d'informations. Elle a, en outre, rendu obligatoire la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. particuliers. Le crédit renouvelable s'inscrivant dans la durée, l'examen triennal de la solvabilité est essentiel : il permet de détecter une éventuelle dégradation de la situation de l'emprunteur. La consultation par le prêteur du fichier des incidents de remboursement ne saurait être le seul outil de détection des situations de fragilité financière, comme le démontrent plusieurs études de la Banque de France sur le surendettement. par la commission spéciale va à l'encontre des préconisations de la Cour des comptes, qui invite au contraire à renforcer l'analyse de la solvabilité des emprunteurs pour le crédit à la consommation.

par des enfants dans des situations difficiles ou des parents qui voient leurs enfants dans des situations difficiles. Quand on voit les pratiques utilisées, avec la possibilité d'emprunter

est à M. le rapporteur. Je souhaite compléter mon propos sur deux points : la lutte contre le surendettement et l'efficacité des mesures législatives. mesures législatives. La lutte contre le surendettement ne repose pas sur la seule vérification triennale de la solvabilité. Le rapport de la Cour des comptes que vous avez évoqué, madame la ministre, préconise d'ailleurs un renforcement de l'analyse de la solvabilité des emprunteurs

effectif. À mon sens, c'est au Gouvernement de prendre ses responsabilités en la matière en proposant les outils nécessaires au contrôle et à la régulation du crédit à la consommation, sans transférer sa responsabilité sur les acteurs du secteur privé. Les professionnels du secteur m'ont indiqué partager l'objectif de lutte contre le surendettement. Simplement, l'obligation de vérification triennale de la solvabilité concerne de moins en moins de contrats de crédit

mesures législatives, j'avoue être un peu déçu par votre position, madame la ministre : oui ou non, cherche-t-on à être efficace collectivement, à simplifier vraiment la vie des entreprises ? Dès lors qu'il s'agit de supprimer des surtranspositions qui représentent un vrai coût pour les entreprises, vous les refusez.

de la compétitivité économique de notre pays. Pour être efficace, mieux vaudrait s'en tenir à des mesures ciblées que de prévoir des mesures systématiques et surtransposées qui,, ne remplissent même pas l'objectif recherché.

il nous paraît particulièrement important de garder ces mesures pédagogiques et intelligibles pour les consommateurs. Comme nous l'avons souligné dans la discussion générale, la responsabilité des entreprises inclut une responsabilité sociale, qui fait partie de leurs missions.

n 6 rectifié et 9 tendent à supprimer l'article 2, que la commission spéciale a approuvé et qui abroge une surtransposition en matière de publicité sur les crédits immobiliers. Plus précisément, cet article supprime l'obligation de mentionner dans les publicités sur les crédits immobiliers trois informations

ces informations sont mentionnées au stade de l'information précontractuelle et contractuelle. C'est d'ailleurs au moment de l'offre contractuelle que l'information est la plus pertinente et la plus utile pour les consommateurs.

des publicités, sans apporter d'informations supplémentaires dont on puisse affirmer qu'elles contribueraient à une meilleure protection du consommateur, qui dispose déjà de toutes ces informations par ailleurs, avant de s'engager contractuellement. Il convient de souligner que la suppression de cette disposition ne remet pas en cause l'existence du délai de réflexion de dix jours : celui-ci est maintenu, et je répète que le consommateur en a nécessairement connaissance avant de contracter, à travers la fiche d'informations qui lui est remise. Par ailleurs, la disposition que supprime le projet de loi fait peser sur le prêteur des obligations de mention qui ne le concernent pas, puisque la subordination de la vente à l'obtention du prêt et le remboursement des sommes versées en cas de refus d'obtention du prêt concernent la relation entre le vendeur et l'acheteur, non la relation entre le prêteur et l'acheteur. Enfin, les mentions dans la publicité qu'il existe un délai de réflexion et que les sommes versées peuvent être remboursées en cas de refus du prêt, si elles sont importantes, ne sont pas vraiment de nature à pousser le consommateur à renoncer à s'endetter en cas de risque d'insolvabilité, de sorte qu'il est difficile d'affirmer que ces dispositions contribueraient à lutter contre le surendettement. Plus généralement,

! Je ne sais pas si, de même que chaque niche fiscale a son chien, chaque surtranposition a son gardien ... En tout cas, je vois que nous aurons beaucoup de mal à arriver à la trentaine de

comprendre qu'elles portaient atteinte aux intérêts des entreprises, il faut renoncer à les simplifier.

aux personnes ce que l'on est en train de leur vendre, je n'accepte pas ! Vraiment, je ne comprends pas votre position

On sait combien il peut pénaliser notre économie, comme il peut être mal compris par les citoyens français. Mais, sincèrement, le texte qui nous est proposé est à la marge. On en reste à l'accessoire, on n'est pas sur l'essentiel. Je suis surpris, madame la ministre, en cet instant, de votre réaction. Effectivement, les sénatrices et les sénateurs ont été privés de la capacité d'enrichir ce texte pour en venir à l'essentiel et vraiment débattre.

Cet amendement porte sur les modalités allégées de publication des comptes des entreprises prévues à l'article 5 du projet de loi. Il apporte plusieurs modifications d'ordre rédactionnel.

c'était le cas avant que la directive n'entre en vigueur - : nous avons un réseau d'avocats, voilà comment il fonctionne et quelles sont ses pratiques. Si vous vous adressez à ce réseau, on paie tout, dans le cas contraire, vous regardez le plafond de couverture, vous payez d'avance et vous serez remboursé une fois la facture reçue. C'était une façon d'inciter les gens à se tourner vers le réseau d'avocats désignés par la compagnie d'assurance. Or le libre choix est fondamental. Les compagnies d'assurance voudraient agir ici comme elles le font en matière de

un procès, l'important c'est pouvoir avoir une relation de confiance entre l'avocat et son client ; celle-ci est fondamentale. Si le libre choix de l'avocat n'est pas garanti, l'assurance de protection juridique devient une compagnie d'assurance qui assure une clause de direction du procès. Lorsque nous avions auditionné à l'époque avec Philippe Bas les compagnies d'assurance à propos de la protection juridique, ces dernières nous expliquaient précisément que leur souhait

cet article supprime l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit. Cette suppression nous dit-on, par le fait que cette interdiction ne serait pas prévue par la directive du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et les articles visés du code des assurances et du code de la mutualité, modifiés par l'article 6 du projet de loi, résultent de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. Le dispositif ainsi mis en oeuvre par le droit interne en 2007 est clairement antérieur à la directive du 25 novembre 2009. Dès lors, il ne saurait y avoir de surtransposition de la directive de 2009 par une loi datant de 2007. Vous l'avez compris, on ne peut pas parler ici de surtransposition. En outre, l'intervention de l'assureur aux côtés de l'assuré pour négocier les honoraires avec son avocat est contraire au principe de libre détermination des honoraires entre l'avocat et son client. Une telle intervention aurait pour conséquence de soumettre la défense de l'assuré à un tarif proposé et, en pratique, imposé par l'assureur. la présence de l'assureur aux côtés de l'assuré lors de la négociation des honoraires de l'avocat peut remettre en cause le libre choix de l'avocat reconnu par la directive. La compagnie d'assurance pourra indiquer à l'assuré que, s'il choisit tel avocat, avec lequel elle a un accord, les honoraires qu'elle acceptera d'avancer seront intégralement pris en charge, ce qui risque de ne pas être cas dans une autre hypothèse. L'assuré sera alors fortement incité à choisir l'avocat ainsi désigné par son assureur, renonçant ainsi à son droit de choisir librement son avocat, ce qui est contraire contraire au principe cardinal consacré par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé que le justiciable ayant souscrit une assurance de protection juridique doit, en toute circonstance, pouvoir décider de l'opportunité de faire appel à l'assistance de tel ou tel avocat, sans que l'assureur lui impose un avocat particulier. Tels sont les arguments essentiels justifiant cet amendement de suppression de l'article 6. La parole

par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de la protection juridique, soit deux ans avant l'adoption de la directive européenne du 25 novembre 2009, dite Solvabilité 2.

entre ce dernier et son client. Comme on le sait, la profession d'avocat est régie par le principe de la libre fixation des honoraires. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « les honoraires [ ...] de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ». Ce principe a été consacré par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que par la Cour de cassation. Aussi, introduire l'intervention de l'assureur dans la négociation des honoraires risque de remettre en cause cette liberté. D'une part, l'assuré se verra proposer des tarifs correspondant au montant de la prise en charge supportée par son assurance. D'autre part, les assureurs pourront former des ententes entre les compagnies sur les prix de leurs prestations de protection juridique, des ententes prohibées par le droit européen. Pour ces raisons, il est souhaitable de laisser en l'état les dispositions prévues par la loi de 2007 précitée.

met fin à l'interdiction faite aux assureurs d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de protection juridique. La commission spéciale a approuvé cet article, qui supprime une surtransposition et que j'estime tout à fait opportun sur le fond. En premier lieu, rien n'imposait de prévoir cette interdiction en droit français. Il s'agit donc d'une surtransposition. En second lieu, j'approuve complètement le dispositif proposé, dont l'objectif est de permettre aux assurés de s'appuyer sur leur assureur dans la négociation avec l'avocat, afin de bénéficier de tarifs plus avantageux. Contrairement à ce que vous avez dit, mon cher collègue, il ne remet pas en cause la liberté pour l'assuré d'un contrat de protection juridique de choisir son avocat, liberté qui constitue, je le rappelle, une prescription européenne, consacrée à l'article L. 127-3 du code des assurances. L'assureur ne pourra toujours pas proposer le nom d'un avocat à son assuré, sans demande écrite de la part de ce dernier. Même dans ce cas, l'assuré sera toujours libre de choisir un autre avocat que celui qui lui est proposé pour l'assister. Enfin, rien n'interdira, lors de la négociation, de convenir, si la complexité de l'affaire le justifie, que les honoraires dépasseront le plafond garanti par l'assureur et que le solde demeurera à la charge de l'assuré, comme c'est le cas actuellement.

Je suis très gêné quand des parlementaires, qui sont avocats ou ont des liens personnels avec un avocat, n'expriment pas publiquement leur potentiel conflit d'intérêts.

En effet, l'interdiction faite aux assureurs de négocier les honoraires directement avec leurs avocats partenaires s'avère pénalisante pour les assurés. Cette interdiction prive les consommateurs d'éventuels tarifs compétitifs pouvant être obtenus par les compagnies d'assurance, faisant usage de leur position d'acheteurs en gros. L'article 6 du projet de loi, qui supprime cette interdiction, est donc favorable aux consommateurs. Cette mesure est d'ailleurs soutenue par les associations de consommateurs, qui ont rencontré la mission inter-inspections. En outre, comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis, et comme l'indique le rapporteur de la commission spéciale, le libre choix de l'avocat, le principe de libre détermination des honoraires et le secret professionnel ne sont nullement remis en cause par cet article, les dispositions garantissant ces principes, tant dans le code des assurances et le code de la mutualité que dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne sont pas modifiées et demeurent applicables. Ainsi, le client assuré sera toujours en droit de recourir soit à un avocat choisi par lui, soit à un avocat proposé à sa demande par sa compagnie d'assurance. De plus, même si l'avocat est proposé par la compagnie d'assurance, l'assuré demeurera libre de négocier les honoraires avec son avocat, indépendamment des accords conclus par ce dernier avec l'assureur et, finalement, de faire part de son accord ou de son désaccord sur le montant des honoraires proposés. il n'existe aucun risque d'atteinte au secret professionnel qui résulterait de la négociation entre les avocats et les assureurs, faisant usage de leur situation d'acheteurs en gros. Ces négociations devront se faire dans le respect du secret professionnel, qui est bien évidemment opposable à l'assureur. Seul l'assuré peut être éventuellement tenu de rendre des comptes à son assurance sur l'évolution de l'affaire et les diligences accomplies, comme cela est déjà le cas actuellement. Enfin, pour répondre à la question de savoir si nous luttons ou non contre une surtransposition, il est exact que la loi était antérieure à la directive, mais nous luttons contre cette forme d'inertie juridique consistant à ne pas adapter notre législation nationale à la directive lorsqu'elle a été adoptée.

vos propos peuvent s'entendre, dans la réalité, dans les faits, cela n'est pas le cas. C'est pourquoi nous voterons ces deux amendements de suppression.

l'assuré demeurera libre d'en choisir un autre ou de négocier les honoraires avec cet avocat indépendamment des accords conclus avec l'assureur. Mais pensez-vous réellement que c'est de cette manière que cela va se passer ? ? Je crois que, dans la vraie vie, ce n'est pas ainsi que cela se passe. L'assuré acceptera la proposition de son assureur avec les travers que j'ai signalés en présentant mon amendement. souvent parce qu'il n'en connaît pas d'autres ou parce qu'il craindra que, s'il n'accepte pas la position de l'assureur, celui-ci, comme cela arrive pour ce qui

lui les germes d'une véritable atteinte au libre choix de l'avocat, ainsi qu'à la libre détermination des honoraires. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

les honoraires d'avocat ne sont pas forcément connus, ils ne sont pas transparents. Certains ordres avaient un temps essayé de donner des mercuriales, mais on s'oppose là aux règles de la concurrence.

Suite du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (procédure accélérée)